a émis un avis favorable, par 21 voix pour et 18 voix contre, à la nomination de M. Philippe Mauguin aux fonctions de président de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 179 au sein de l’article 3.

aussi des objectifs plus généraux tels que la fermeture du cycle du combustible nucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle de l’hydrogène bas carbone.

à renforcer le soutien apporté au développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides, refroidis au sodium, et à la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel de la filière. Il s’agit ici de respecter l’esprit des conclusions de la commission d’enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050.

Les risques de dissémination nucléaire sont réels. Par ailleurs, pour ce type de nouvelle technologie, les questions de gestion de la sûreté, d’une part, et de gestion de la sécurité des sites, d’autre part, sont fondamentales. Quels sont les moyens pour assumer ces missions sur les sites d’implantation ?

la stratégie française pour l’énergie et le climat prévoient de développer un petit réacteur modulaire et un petit réacteur innovant dès 2030. D’autre part, l’amendement semble déjà satisfait. En effet, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) qui, en tant qu’autorité administrative indépendante,

le mix énergétique dépend des contraintes techniques et industrielles. Eu égard aux contraintes industrielles et de sûreté nucléaire, il ne peut être exclu que la part du nucléaire en 2050 soit légèrement inférieure à 50

Le scrutin est ouvert.

L’amendement n° 149 est présenté par le Gouvernement.

Les travaux relatifs aux 8 réacteurs supplémentaires sont en cours. À mon sens, il importe d’éviter de figer prématurément la puissance totale et le nombre de réacteurs qui seront construits à l’horizon 2050, afin de se préserver une latitude suffisante en matière d’innovation et de diversité des projets. Il convient aussi, selon moi, de ne pas s’enfermer dans une technologie : on étudie la possibilité de construire 6 réacteurs supplémentaires,

À l’inverse, adopter l’amendement n° 134 éroderait l’ambition initiale de l’article 3. La rédaction suggérée ne permettrait de cranter que la construction de 23 gigawatts d’ici à 2030, correspondant aux 14 EPR2 et à un premier SMR. J’ajoute que mentionner maîtrise publique poserait une difficulté au regard des règles de la commande publique. Au reste, elle n’est pas nécessaire, puisque la loi Nouveau Nucléaire du 22 juin 2023, qui doit servir de socle à la relance du nucléaire, ne permet la construction d’EPR2 que dans les sites existants déjà nucléarisés,

Yannick Jadot, pour explication de vote. Je voudrais abonder dans le sens de mes collègues. EDF fait déjà face à un mur d’investissement absolument colossal

à engranger des profits avec de plus en plus de mégawattheures négatifs, d’autant que les autres pays avancent à marche forcée sur les énergies

Merci,

Sur cet amendement,

Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à adapter la rédaction de l’article en retenant un objectif de disponibilité des installations nécessaires au traitement et au recyclage des combustibles nucléaires usés.

particulièrement stable, en vue de leur stockage. Le dernier conseil de politique nucléaire a validé le lancement d’un programme d’ampleur visant à poursuivre au delà de 2040 la stratégie française pour l’aval du cycle du combustible. Il semble indispensable que ce programme d’ampleur soit mené par Orano en tenant compte des impératifs de gestion durable des substances radioactives. Il conviendra notamment que les filières nucléaires examinent les innovations à prendre en compte dans une logique de préparation de la fermeture du cycle de sécurité d’approvisionnement. Il importera qu’Orano mène ce programme en évitant toute interruption de service qui affecterait le parc électronucléaire d’EDF. Orano doit également tenir compte de la maîtrise des coûts. Il faut enfin que le schéma de financement et de gouvernance de l’aval du cycle du combustible comporte les incitations nécessaires à son succès.

Mme la ministre déléguée. Si le Gouvernement partage l’objectif de tendre vers la fermeture du cycle du combustible, la proportion de matières recyclées pour le fonctionnement des réacteurs nucléaires relève d’une optimisation économique et industrielle à laquelle il convient de laisser une latitude suffisante, au bénéfice de l’efficacité d’ensemble. Cette optimisation peut, par exemple, conduire à prendre en compte la situation du marché de l’uranium ou à conserver des matières en vue d’une consommation ultérieure dans des réacteurs de quatrième génération.

de capacité de flexibilité électrique et de captage de dioxyde de carbone. Monsieur Jadot, vous voulez non pas du nucléaire, mais des énergies renouvelables. Mais il faut aussi garantir la stabilité du réseau. C’est pourquoi le Gouvernement estime nécessaire de procéder à des développements ambitieux dans ce domaine, même s’il convient d’être prudent dans la fixation d’objectifs quantitatifs et de prendre en compte les moyens de flexibilité de manière plus intégrée que ne le prévoit l’article 4. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement

Vincent Delahaye, vise à promouvoir les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, en laissant inchangés la propriété publique et l’équilibre financier des réseaux publics de distribution d’énergie.

d’introduire de la planification territoriale énergétique et de tenir compte des spécificités et contraintes de chaque territoire, tout en garantissant une juste répartition de l’effort de réduction de l’empreinte carbone sur l’ensemble du territoire.

en matière d’énergie et de climat. Ensuite, il y a des modalités de répartition de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ce sont les États, et non les collectivités ou les entreprises, qui sont parties à l’accord de Paris En application de cet accord, les États doivent ainsi soumettre des contributions déterminées au niveau national (CDN). C’est à cette échelle que doit juridiquement s’apprécier l’effort des États dans la lutte contre le changement climatique.

la territorialisation des objectifs de réduction des émissions risquerait de provoquer un débat stérile, qui croise à des logiques de responsabilités communes, mais différenciées, souvent bloquantes.

est important que les COP régionales, au travers des comités régionaux de l’énergie, puissent décliner les quantités à produire et que les territoires aient le droit de choisir ce qui leur paraît le plus opportun et le moins dégradant pour l’environnement : avoir 2 000 éoliennes sur le territoire départemental de la Somme, c’est insupportable

L’autoconsommation d’électricité constitue un moyen efficace pour accélérer la transition écologique et sécuriser l’approvisionnement énergétique. Elle s’inscrit donc pleinement dans la stratégie française visant à améliorer la résilience du mix énergétique.

Cet amendement vise à faire du développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment collective, un pilier de la politique énergétique et climatique française, en rattrapant le retard sur nos voisins européens et en menant une action pour lever les freins, notamment réglementaires et fiscaux.

produit à partir de gaz naturel, afin d’atteindre l’objectif de 77 % d’utilisation d’hydrogène propre dans l’industrie en 2030. Quel est l’avis de la commission ?

d’hydrogène uniquement renouvelable dans la consommation d’hydrogène relative en 2030 et 48 % en 2035. Cette voie est ouverte si l’objectif d’énergie renouvelable dans le mix électrique est atteint 44 % en 2030 – et si la part de l’hydrogène électrolyte renouvelable ou bas carbone ou de ses dérivés utilisés dépasse en France 77 % en 2030 et 80 % en 2035. Voilà rappelés tous les objectifs. La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit bien le second cas ouvert par la directive nous permettant de bénéficier de notre électricité bas carbone. Je vous propose de nous en tenir à la rédaction actuelle. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

amendement vise à étendre l’objectif de développement du stockage pour formuler un objectif plus global portant sur l’ensemble des flexibilités de la modulation de la consommation et du stockage, dans le respect de la neutralité technologique. Cette proposition est cohérente avec les conclusions de la commission d’enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050. Elle l’est également avec la réforme du marché européen de l’électricité.

de stockage de CO2 peut être pertinente dans un certain nombre de cas, notamment pour certains secteurs industriels, mais qu’elle ne peut nullement être exonératoire pour l’ensemble des producteurs de gaz carbonique. Il n’est pas question, passez moi l’expression, de monter des usines à gaz partout en s’exonérant de toute autre solution de

La technologie de captage, utilisation et stockage de CO2 ne constitue aujourd’hui qu’une piste de recherche parmi les nombreuses solutions de décarbonation de notre économie. Lors du Conseil national de l’industrie, au mois de juin 2023, le gouvernement a annoncé le lancement d’une consultation publique sur un projet de stratégie de captage, stockage et utilisation de CO2. Plus largement, la question de ce recours fait l’objet de débats parmi les acteurs économiques. Certains acteurs plaident pour l’utiliser davantage ; à l’inverse, d’autres appellent à cibler son utilisation sur la décarbonation de l’industrie plutôt que la production d’hydrogène. De nombreuses questions, voire contradictions, ont été soulevées sur ce point dans le rapport sénatorial d’information sur la décarbonation des transports du mois de juillet dernier. Comment se fixer des objectifs chiffrés sans avoir au préalable mené un rapport sérieux et complet ?

recours annuel à ces technologies d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050. Ces nouvelles technologies, qui consistent à capturer le dioxyde de carbone produit par divers processus industriels, à le transporter, puis à le stocker sous la terre ou sous la mer, suscitent un intérêt et un engouement croissants, notamment du fait de l’accroissement de la valeur financière de la tonne de carbone. Pour autant, ces technologies n’ont à cette date fait la preuve ni de leur fiabilité ni de leur efficacité. Les coûts de ces infrastructures, non seulement de captage et de stockage, mais aussi de transport, restent très élevés, alors que les bénéfices attendus demeurent incertains, ces incertains, ces technologies n’étant pas encore matures. En outre, force est de souligner que le bilan carbone de ces technologies demeure controversé. Elles sont, en effet, fortement consommatrices d’énergie, et le transport du CO2 capté nécessitera quant à lui la création de centaines de kilomètres de canalisations supplémentaires. Il s’agit donc de compléter cet alinéa en précisant que le recours à ces technologies ne peut être considéré comme un substitut aux efforts de décarbonation que doivent réaliser les secteurs d’activité fortement émetteurs de CO2. Quel

émet donc un avis défavorable.

en cohérence avec l’amendement n° 158. Il s’agit de privilégier le principe d’un objectif global qui porte sur l’ensemble des flexibilités, dans le respect de la neutralité technologique. Cette proposition est cohérente avec les conclusions de la commission d’enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050. Elle l’est également avec la réforme du marché européen de l’électricité. Selon les travaux de RTE dans son rapport, le système électrique nécessitera entre

Cette mission a mis en évidence les enjeux liés à la concurrence des usages des biocarburants, s’agissant tant de la disponibilité des matières premières utilisées pour fabriquer ces carburants, en particulier la biomasse, que de leur meilleure utilisation possible au regard de leur rendement et des alternatives pour contribuer à la décarbonation de tel ou tel secteur. Nous souhaitons renforcer le suivi des ressources de biomasse au travers d’instances, de schémas nationaux permettant d’élaborer

Madame la ministre la PPE actuelle ne fixe pas d’objectifs chiffrés pour l’hydrolien, mais la future PPE pourra prévoir le lancement de premiers appels d’offres commerciaux sur l’hydrolien, sous réserve de l’évolution des coûts de la technologie.

À un moment donné, il faut avoir une vraie volonté politique pour mettre en place les hydroliennes que nous attendons, notamment dans l’ouest de la France, où nous avons de très forts courants.

100 4 du code de l’énergie par un nouvel objectif : mobiliser davantage la biomasse énergétique en faisant de la sécurité alimentaire, de la préservation de la biodiversité et du potentiel de stockage de carbone forestier

s’articuleraient mal avec ce droit existant. En effet, l’objectif ferait référence à la stratégie nationale bas carbone mentionnée à l’article L. 222 1

amendement ne respecteraient pas le principe de neutralité technologique. En effet, les granulés de bois seraient la seule technologie à laquelle il serait explicitement prévu

à charbon. La production d’électricité à partir de biomasse ne pourra être développée que sous conditions, notamment en soutien d’activités industrielles. Cette activité ne constitue pas une priorité d’usage de la biomasse. Elle devra être examinée

M. Gilbert Luc Devinaz. Cet amendement vise à intégrer la question fondamentale de la préservation de la ressource en eau dans un contexte de réchauffement climatique et de conflits d’usage potentiels. En effet, qu’il s’agisse de la production hydroélectrique, du refroidissement des centrales nucléaires, de la production sylvicole et agricole pour la biomasse ou d’autres ressources mobilisant d’importantes quantités d’eau pour la production d’énergie ou de chaleur ou dans le cadre des process liés à la fabrication des équipements nécessaires à ces installations de production, l’accélération du changement climatique est un enjeu majeur pour notre gestion de la ressource en eau.

par la loi Énergie climat du 8 novembre 2019 –, ne mentionne quasiment pas l’articulation des activités de production d’énergie avec les effets du changement climatique. C’est une regrettable omission imputable à l’obsolescence de ce titre, qu’il convient donc de corriger. la rédaction de cet amendement me semble suffisamment souple pour ne pas entraîner de difficultés pour les centrales hydroélectriques ou nucléaires. En effet, elle précise que cet objectif doit être poursuivi « sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ». Pour ces raisons, madame la ministre,

Quel est l’avis de la commission ? La modification proposée ne me semble pas souhaitable. Les carburants de synthèse étant une technologie très neuve, il est prématuré de fixer un objectif contraignant dans le secteur du transport maritime.

M. Gilbert Luc Devinaz. Afin d’atteindre les objectifs de décarbonation du secteur des transports notamment, il est indispensable de raisonner en termes de bilan carbone et d’efficacité énergétique, plutôt qu’en termes technologiques.

À titre d’illustration, l’article L. 100 4 du code de l’énergie fait référence à « environ 7 % » en 2023 en ce qui concerne la réduction de la consommation totale.

qu’ils sont portés par les exploiteurs des centrales. En effet, les projets de reconversion de centrales à charbon vers des combustibles bas carbone sont des projets à long terme, qui suivent généralement des calendriers de plusieurs années.

du Gouvernement ? Cette précision rédactionnelle ne semble pas de nature à clarifier le texte. En effet, des projets de reconversion peuvent, le cas échéant, être portés par d’autres acteurs que l’exploitant. Par ailleurs, la rédaction proposée reste imprécise. Les termes « sous réserve des projets de reconversion » laissent entendre que l’interdiction ne s’applique que sous réserve de la mise en œuvre de ces projets, alors que le sens recherché est que l’interdiction s’applique « sauf pour ces projets ». Pour ces raisons, le

de leur éradication une priorité. La précarité énergétique s’accroît, et le nombre de logements qualifiés de passoires thermiques ne baisse pas, car trop peu de personnes s’engagent dans un parcours de rénovation. Plus de la moitié des passoires thermiques sont pourtant des maisons individuelles, mais seulement 32 % du parc privé ont fait l’objet de travaux de réhabilitation. La raison de cette près de la moitié des ménages résidant en passoire thermique a des revenus modestes, voire très modestes – 37 % de ces logements sont occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il est nécessaire de recentrer l’effort budgétaire du pays sur les passoires thermiques, afin de sortir 5,6 millions de ménages de la précarité, qu’ils soient propriétaires ou copropriétaires, bailleurs ou occupants. Dans cette perspective et dans un souci de pragmatisme, il est également proposé de permettre au propriétaire occupant de réaliser les travaux de rénovation globale en plusieurs tranches, financé et accompagné et dans un délai inférieur à six ans à compter du début d’exécution des travaux, à condition que ces derniers soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. le délai actuel de dix huit mois nécessite souvent un relogement et ne permet pas d’étaler les paiements dans le temps. Quel est l’avis de la commission ? Ces amendements de la commission ? Ces amendements tendent à modifier, dans des sens différents, les objectifs afférents à la rénovation énergétique. L’amendement n° 36 vise à rénover prioritairement les passoires thermiques et à modifier la définition de la rénovation énergétique globale.

Or c’est sur l’État, non sur ces collectivités, que doit reposer prioritairement l’effort public en matière de rénovation énergétique. Par ailleurs, la définition de moyens budgétaires relève davantage d’une loi de finances que de la présente proposition de loi de programmation et de simplification. Quel un avis défavorable

au réseau métropolitain continental l’objectif de tendre vers l’autonomie énergétique à l’horizon 2050. En premier lieu, nous estimons qu’il est nécessaire de fixer comme objectif programmatique celui d’atteindre cette autonomie en 2050.

fixés : à l’horizon 2030, un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables ; à l’horizon 2050, l’autonomie énergétique. Comme l’a souligné le groupe de travail

comme l’Hexagone, que soit formalisé pour chacune d’elles un document d’orientation et de programmation stratégique spécifique fixant à ces territoires

à l’horizon 2030 et de mix énergétique autonome à l’horizon 2050 dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les ZNI.

au premier rang desquels les énergies de récupération, qui doivent pouvoir trouver toute leur place dans les objectifs de la politique énergétique. La valorisation énergétique des déchets, la récupération de la chaleur fatale générée par les sites industriels, les ou encore le traitement des eaux usées sont autant de leviers qui contribuent à transformer les ressources locales de nos territoires en une énergie locale décarbonée. Les énergies de récupération doivent donc pouvoir trouver toute leur place dans la politique énergétique et dans la réponse à apporter en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En effet, il vise à ajouter les énergies de récupération aux côtés des énergies renouvelables dans l’objectif de mix renouvelable à l’horizon 2030 dans les zones non interconnectées au réseau, les ZNI.

La loi européenne sur le climat fait de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 une obligation légale. Alors que nous blâmons régulièrement le Gouvernement de surtransposer le droit communautaire, il ne s’agirait pas de nous placer désormais à rebours du droit européen.

Nous sommes d’accord : la diminution de la captation du carbone par la forêt pose un problème de taille pour atteindre nos objectifs climatiques. La stratégie nationale bas carbone, élaborée en 2018 2019, mise sur une hausse de la capacité de stockage des forêts d’ici à 2050 pour parvenir à la neutralité carbone à cette date, comme nous nous y sommes engagés.

de respecter nos obligations européennes. Pour rappel, selon les scientifiques, si l’on veut rester dans le cadre de l’accord de Paris, il faudrait que l’Europe atteigne la neutralité carbone en 2040 et que l’objectif pour 2030 soit de 65 % de réduction.

Je rappelle que la rédaction retenue, à savoir « tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre en excluant les émissions et les absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie de 50 % d’ici 2030 », est issue de l’article 1 de l’avant projet de loi sur la souveraineté énergétique. Par ailleurs, cette même rédaction figure dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans la stratégie française pour l’énergie et le climat.

Les résultats des politiques publiques en la matière sont peu quantifiables sur des laps de temps très courts. Notre boussole doit donc rester, pour les émissions nettes, l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050. Par ailleurs, nous ne serons fixés sur le véritable objectif de la France

terre à terre sur le sujet et encourageons le développement de ce biogaz.

qui ne me semble pas souhaitable. Nous avons déjà défini un objectif en faveur des solutions pour les foyers ruraux non raccordés aux réseaux d’électricité, de gaz ou de chaleur au 2° de l’article L. 100 2 du code de l’énergie

Merci,